La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 13 mai 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Michel Souplet, qui fut sénateur de l'Oise de 1983 à 2001, et de Roland Povinelli, qui fut sénateur des Bouches-du-Rhône de 2008 à 2014. avons terminé avec le débat sur les perspectives de la saison estivale, notamment pour les activités touristiques et culturelles, au regard de la situation liée à l'épidémie. 364, avis n° 363). Mes chers collègues, notre séance se déroule dans les conditions de respect des règles sanitaires mises en place depuis le mois de mars. L'hémicycle fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection avant et après chaque séance. Les micros seront désinfectés après chaque intervention. J'invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité. Je rappelle également que les sorties de la salle des séances devront exclusivement s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle. de l'hémicycle. Tous les orateurs, y compris les membres du Gouvernement, s'exprimeront depuis leur place, sans monter à la tribune. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

veux rendre hommage aux professionnels du tourisme, à ces deux millions d'hommes et de femmes qui font fonctionner les hôtels- petits et grands -, les maisons d'hôtes, les résidences de tourisme, les campings, les restaurants, les villages de vacances, les centres de congrès, les salons, les musées,

Ensemble, ils créent 7 % à 8 % de la richesse nationale chaque année. Ils attirent 90 millions de touristes et participent ainsi au rayonnement de notre pays dans le monde entier. Aujourd'hui, je veux leur témoigner tout mon soutien. Le secteur du tourisme est probablement le plus durement touché par cette crise hors du commun qui a mis à l'arrêt notre pays du jour au lendemain. Il avait toutefois déjà été touché, dès le début de l'année, par la diminution du trafic international de voyageurs et, encore un peu avant,

des innombrables compétences et savoir-faire qui sont les nôtres et que le monde entier nous envie. Le bilan du premier semestre est terrifiant, et le retour à la normale ne pourrait avoir lieu qu'en 2022. Il faut le souligner, monsieur le secrétaire d'État, l'État s'est pleinement mobilisé pour tenter d'apporter une réponse adéquate à la crise. Des mesures spécifiques ont été annoncées les 24 avril et 14 mai derniers.

Les professionnels attendent également des gestes quant aux loyers du parc privé, dans la logique « zéro recette, zéro charge ». Le chômage partiel pourrait être élargi à certains professionnels dont les effectifs n'ont été mobilisés que pour gérer les pertes

Les plateformes en ligne devraient être appelées à témoigner de leur solidarité envers leurs partenaires les plus fragiles, à travers une diminution temporaire des commissions. viens aux mesures de nature à favoriser la reprise. Les droits au chômage des saisonniers devront être élargis afin de faciliter leur embauche pour la saison estivale. Une garantie d'État exceptionnelle des avoirs proposés par les hébergeurs et par les compagnies aériennes pourrait être mise en place, pour réinstaurer la confiance des consommateurs. Il est également urgent de légiférer à l'échelon européen sur les avoirs proposés par les compagnies aériennes. Enfin, pour relancer le tourisme à moyen terme, la prochaine génération de contrats de plan État-région devrait être utilisée pour financer des appels à projets visant à mieux répartir les flux touristiques sur notre territoire, qui souffre de la fameuse règle des 80-20, que l'on connaît dans d'autres domaines.

-est celle du périmètre concret de ce que le Gouvernement appelle le tourisme. En effet, de nombreux professionnels restent dans le flou. Je pense aux entreprises qui approvisionnent les cafés, restaurants et toutes les manifestations culturelles et sportives, comme les grossistes en boissons, aux blanchisseries, aux conciergeries pour les meublés de tourisme, aux agences immobilières spécialisées dans la location de meublés, à l'agritourisme, et j'en passe. Concernant Concernant l'événementiel, je signale une ambiguïté dans le dossier de presse publié dans la foulée du comité interministériel du tourisme (CIT), à laquelle il faut remédier : le détail des mesures n'évoque que « l'événementiel culturel et sportif », excluant ainsi l'événementiel d'affaires ou privé, ce qui n'est évidemment pas souhaitable.

les professionnels craignent par-dessus tout de se retrouver face à un « mur » en cas de levée soudaine et générale de ces mesures une fois l'activité reprise. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous les rassurer sur le fait que ces mesures accompagneront la reprise et ne diminueront que de façon progressive ?

Par ailleurs, je regrette que rien n'ait encore été décidé pour le tourisme social, si cher, à juste titre, à notre collègue Viviane Artigalas, ni pour la solvabilisation de la demande pour cet été. La cellule « Tourisme » de la commission des affaires économiques a préconisé la mise en place d'un dispositif exceptionnel d'aide au départ en vacances s'appuyant sur les chèques-vacances, une diminution exceptionnelle des tarifs autoroutiers cet été et des dispositifs d'aide pour certains publics ciblés. Nous devons faire en sorte que les Français partent en vacances ! Le tourisme domestique représente les deux tiers des recettes du secteur. En capitalisant sur cet atout, nous pouvons limiter la casse. un mot sur les allégements de fiscalité locale. L'État s'est engagé à prendre en charge la moitié de l'exonération de la CFE pour les collectivités qui le décideraient.

je formulerai une remarque d'ordre général. La politique du tourisme en France comme son budget ne cessent de s'amenuiser depuis de nombreuses années, en raison du sentiment erroné selon lequel « le tourisme fonctionne tout seul alors qu'il s'agit d'une économie diffuse qui a besoin de l'action de l'État et des différentes collectivités, en particulier des communes, pour créer la synergie nécessaire à cette bioéconomie.

Elle démontre à nouveau la nécessité de nommer un ministre du tourisme de plein exercice, qui s'appuierait sur une direction d'administration centrale dédiée. Monsieur le secrétaire d'État, soyez assuré que nous serons vigilants quant à la bonne application du plan Tourisme sur nos territoires.

de recettes. C'est colossal ! C'est pourquoi, dès le 24 avril, le Président de la République, recevant un certain nombre de représentants du secteur, notamment le bureau du comité de filière tourisme, a appelé à faire du tourisme une priorité nationale et a déclenché la préparation d'un plan de sauvetage, qui s'est traduit, la semaine dernière, lors du CIT, par l'annonce de dispositifs non seulement de soutien

Ce plan de sauvetage massif permet de donner de la visibilité à un certain nombre de dispositifs : l'activité partielle et le fonds de solidarité se poursuivront jusqu'à la fin de l'année 2020,

Je veux d'ores et déjà rassurer un certain nombre de secteurs. Nous avons fait en sorte que des secteurs qui sont annexes ou connexes, mais qui dépendent parfois de façon importante du secteur du tourisme, puissent bénéficier de ces exonérations, dès lors que ces structures peuvent prouver une perte de chiffre d'affaires significative. C'est le cas pour les grossistes en boissons ; ce sera le cas pour la blanchisserie qui est liée à ce secteur

un travail de dentellière et que nous essayons de raccrocher au maximum tous les acteurs économiques qui nous signalent subir l'impact de cette crise économique

d'une sorte de déclic psychologique : depuis jeudi, les demandes d'information et les réservations augmentent de façon significative ; tous peuvent en attester.

du travail au comité de filière, avec tous les territoires, d'ici à la fin de l'année, avec un point d'étape au mois de juillet. Je crois qu'il est important de mettre toutes nos forces pour que la France reste la première destination, même s'il faut une répartition harmonieuse des flux- je reprends

une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

Avec presque 90 millions de visiteurs étrangers pour la seule année 2018, la France est aussi le pays le plus visité du monde. Son tourisme est grandement culturel. Son patrimoine, d'une richesse incomparable,

Parmi ces monuments historiques, 44 % sont des propriétés privées, soit des biens familiaux, soit des biens acquis par des passionnés. Derrière la carte postale architecturale se cachent des entrepreneurs, des PME parfois, qui se battent pour faire vivre leur passion : 90 % de leurs recettes proviennent souvent de la billetterie, donc des visites et du tourisme. Ces merveilles du patrimoine français ont besoin d'être restaurées et entretenues en permanence. Ces sites sont également synonymes d'emplois et de savoir-faire très divers où plusieurs corps de métier se croisent, des permanents tout comme des saisonniers. un exemple parmi tant d'autres. Dans mon département, la Seine-et-Marne, la famille de Vogüé, propriétaire du prestigieux château de Vaux-le-Vicomte, a dû en fermer les portes et mettre, depuis de ses salariés au chômage technique. Pourtant, il faut continuer à entretenir le domaine, et les charges incompressibles courent.

Les visiteurs étrangers seront beaucoup plus rares, mais la crainte de partir à l'étranger peut bénéficier au tourisme national. Comme le dit si bien Stéphane Bern, « le patrimoine est une passion française

Une partie de l'offre est de nouveau accessible, au terme d'un dialogue entre préfet et élus, et c'est tant mieux. Quoi qu'il en soit, on sait combien ce patrimoine est lourd à entretenir. C'est pourquoi les entreprises de gestion de monuments historiques font partie du périmètre des entreprises qui pourront bénéficier

portée par Atout France est dotée de 21 millions d'euros- c'est considérable, c'est beaucoup plus que ce que nous avions jusqu'à maintenant. Ce sera un soutien précieux. Par ailleurs, les initiatives parlementaires ont été

les deux tiers de la cotisation foncière des entreprises de tourisme, l'État en finançant la moitié. Si les collectivités locales, comme les professionnels, se réjouissent de ce plan, beaucoup s'interrogent néanmoins sur ses dispositions précises. En effet, la taxe de séjour n'a jamais été identifiée comme un élément déclencheur de séjour des touristes : on ne choisit pas sa destination en fonction du montant de la taxe de séjour. Par ailleurs, celle-ci est financée par le touriste et non par

En revanche, c'est synonyme d'une perte nette de recettes pour des collectivités qui en sont déjà privées depuis plusieurs mois et qui doivent assurer, là, la promotion, là, le salaire des agents, parfois même des offres touristiques pour lesquelles elles ne connaissent pas encore à ce jour les protocoles sanitaires, donc les surcoûts.

comment ils s'équilibreront. Les collectivités locales chargées du tourisme ont pour habitude d'adapter au plus juste leurs taxes, en fonction des réalités et des politiques touristiques. Leur demander de diminuer leurs recettes, c'est les mettre en difficulté face à ces enjeux majeurs dont nous parlons, c'est fragiliser leurs capacités à assumer le rôle de levier que nous leur demandons tous pourtant de tenir. Et que dire des départements et de leurs agences de développement touristique, amputées de la taxe supplémentaire additionnelle- 10 % de la taxe de séjour ? Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous expliquer en quoi diminuer les marges de manoeuvre financières des collectivités locales gestionnaires des compétences touristiques est une option à la fois nécessaire et réaliste pour prendre le virage de la relance, des innovations et de la transformation, attendu dans les territoires ?

Dans un tel scénario, c'est une part bien plus grande du PIB qui serait en danger. Mon département, la Haute-Savoie, est le deuxième département le plus touristique de France. En l'absence de mesures fortes pour aider le tourisme des quatre saisons- lacs et montagnes -à surmonter cette crise, c'est l'ensemble du système économique du département qui pourrait s'effondrer. Les secteurs que je viens de citer sont intimement liés et interdépendants les uns des autres. L'absence de soutien à l'un entraînerait la faillite de l'autre. À quoi bon partir en vacances si aucune des activités habituellement disponibles en cette période n'est possible ? Je pense aux visites de musées, aux festivals, aux sorties au restaurant- beaucoup de restaurateurs nous indiquent que, suivant les mesures, ils ne sont pas près de rouvrir achats d'articles locaux. Comment partir en vacances si les sociétés de transport ne survivent pas ? Si la mobilisation de près de 18 milliards d'euros par le Gouvernement pour soutenir le secteur touristique est plus que souhaitable, les secteurs qui y sont liés ne doivent absolument pas être oubliés. Il y va de leur survie. L'augmentation L'augmentation du plafond des tickets restaurant pour le secteur de la restauration est déjà un premier pas satisfaisant, mais quelles autres mesures seront prévues pour les secteurs liés au tourisme ? La prolongation du chômage partiel et du fonds de solidarité n'est pas suffisante. Les entreprises de ces secteurs seront déjà victorieuses si elles réalisent ne serait-ce que 50 % de leur chiffre d'affaires habituel. Comment pourront-elles survivre dans ces conditions, tout en finançant la mise en place des mesures de sécurité ? Elles ont déjà engagé des sommes correspondant à quelques milliers d'euros pour assurer le respect des gestes barrières. Ces dépenses devront être renouvelées chaque mois jusqu'à la fin de l'épidémie. Cela n'est pas viable sur le long terme. Ne serait-il pas envisageable de prendre au moins en partie en charge

Le 13 avril, le Président de la République a annoncé la mise en oeuvre de plans spécifiques de soutien de grande ampleur pour les secteurs durablement atteints. Je suis très heureux

culture et tourisme sont fortement imbriqués. Il n'y a pas de tourisme sans culture, comme il n'y a pas de culture sans tourisme. Car donner à voir, c'est donner à voir

sa première intervention dans l'hémicycle. Je tiens tout d'abord à remercier mes collègues pour l'organisation de ce débat. Il nous permet de réfléchir à la sortie de crise et aux modèles de développement que nous souhaitons privilégier dans les mois et années à venir. Mes questions cibleront principalement le tourisme dans les zones rurales et hyper-rurales. Dans mon département, en Lozère, nous avons la chance de bénéficier de deux parcs exceptionnels : le parc national des Cévennes, qui appartient au patrimoine mondial de l'Unesco, et le parc naturel régional de l'Aubrac, plus récent, où se pratique un agropastoralisme fort. Ces parcs offrent, dans l'imaginaire collectif, une carte postale d'un temps presque oublié. Pourtant, tout cela ne s'est pas fait tout seul. À la fin des années 1960, le sous-préfet de Florac, M. Mazerot, avait proposé aux éleveurs des Cévennes des conventions, appelées « contrats Mazerot qui permettaient de rémunérer les éleveurs et les agriculteurs pour des tâches d'entretien de l'environnement, qu'il s'agisse de murets, de terrasses ou de canaux d'irrigation. Monsieur le secrétaire d'État, ces zones naturelles ont aujourd'hui besoin d'aide pour opérer un saut qualitatif important pour les infrastructures d'accueil de touristes. Cet été, les établissements tels que les hôtels, les campings ou les gîtes chercheront à fidéliser une clientèle nouvelle. Un soutien des investissements permettant leur rénovation sera donc indispensable. Compte tenu de leur implantation dans des zones naturelles remarquables, il est évident que ces travaux doivent leur permettre de se conformer aux exigences du tourisme durable et résilient. C'est pourquoi je souhaiterais savoir si le Gouvernement prévoit de travailler à des conventions du type « contrats Mazerot », pour relancer les investissements dans le tourisme vert, particulièrement dans les parcs nationaux et régionaux. régionaux. Enfin, avec la perspective d'un tourisme exclusivement national, voire européen si les conditions sanitaires le permettent, des travaux d'adaptation ainsi que le recrutement de nouveaux saisonniers seront nécessaires dans ces parcs, ce qui pourrait entraîner des dépenses non prévues au budget 2020. Le Gouvernement entend-il mettre en place des aides à cet effet ?

inédite témoigne de l'immarcescible volonté qui anime le Gouvernement de faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Cela étant dit, les perspectives estivales touristiques, ce sont aussi, vous le savez, les quelque 1 200 musées français qui accueillent toute l'année nos concitoyens et les touristes étrangers. Ces musées, qui font le prestige de la France, fonctionnent grâce aux femmes et aux hommes qui y travaillent. Parmi eux se trouvent les guides-conférenciers, aujourd'hui touchés de plein fouet par la crise. Ils sont près de 10 000 à rendre les oeuvres accessibles au public. Par leur truchement, c'est bien la divulgation des oeuvres et l'exception culturelle française qui Reste que les guides-conférenciers sont une population très précaire. En 2019, la succession des mouvements sociaux les a déjà fragilisés en rendant difficile l'accès aux musées. Aujourd'hui, toutes leurs commandes sont annulées. Toutes les salles de conférence et la plupart des musées et sites touristiques sont fermés. Les guides-conférenciers se trouvent, de fait, dans l'impossibilité de télétravailler et sans accès à leur lieu de travail. Si nombre d'entre eux ont le statut de travailleur indépendant et sont donc éligibles au fonds de solidarité, 36 % sont salariés. Ceux qui sont en contrat court, en fin de mission ou en fin de droits ne peuvent toucher ni le chômage partiel ni les 1 500 euros d'aide aux indépendants. Monsieur le secrétaire d'État, qu'est-il prévu pour ces salariés non couverts ? Par ailleurs, l'annonce anticipée de la réouverture des petits musées est tout à fait opportune ; celle des grands musées, à partir du 15 juillet, l'est également. Néanmoins, les groupes de visiteurs, dont l'activité des guides-conférenciers dépend entièrement, seront-ils autorisés dans les musées à partir du 15 juillet ?

que le CIT acte le principe d'un travail sur le traitement des situations particulières des guides-conférenciers salariés privés d'emploi du fait de la crise sanitaire. Nous sommes donc engagés dans ce travail. Par ailleurs, ceux qui sont indépendants peuvent prétendre au fonds de solidarité nationale, avec un premier étage à 1 500 euros et un deuxième étage jusqu'à 10 000 euros, afin de répondre aux situations les plus critiques. Dans certains cas, ils peuvent être éligibles à un PGE, un prêt garanti par l'État. Au demeurant, la réouverture progressive des sites et des monuments sera la vraie réponse.

tout le monde veut désormais visiter notre belle région, ce que je comprends. Le tourisme en PACA, c'est 10 % du PIB, 10 % de l'emploi, 20 milliards d'euros de recettes et 30 millions de visiteurs. Ce n'est pas un secteur important pour l'emploi et l'économie de Provence, c'est vital ! Aujourd'hui, il est en danger de mort : 80 % du personnel hôtelier est en chômage partiel, et ce secteur évalue déjà sa perte de chiffre d'affaires à 40 %. Ces dernières semaines, nos esprits sont restés confinés entre les murs de vos informations contradictoires. On ne suit plus votre logique ; il y a des lieux fermés, comme les supermarchés, qui sont ouverts au public, et des lieux ouverts, comme les forêts, les montagnes et les plages, qui sont fermés au public. Si j'étais taquin ou éclairé, je pourrais en conclure que les hauts lieux du consumérisme, grands pourvoyeurs de TVA, peuvent ouvrir leurs portes, tandis que les lieux de liberté et de ressourcement, où l'on pratique des activités non lucratives, doivent rester Le message est clair : le si bien nommé supermarché a la priorité sur le petit restaurateur de quartier. Envolées déjà les promesses d'un « monde d'après », les intérêts du marché mondialisé priment encore et toujours sur l'économie réelle. Maintenant que s'approche la période estivale, il faut entendre les deux besoins qui pressent. rendre la liberté d'aller et venir, de s'épanouir, quels que soient les lieux, afin que chacun reprenne possession des chemins, des bars, des restaurants et des rues. Ensuite, il est nécessaire de rendre la liberté d'entreprendre, de travailler, de recevoir ses clients et de remplir les carnets de commandes. Il faut de toute urgence annuler les charges sociales et fiscales des entreprises de la filière touristique, qui ont perdu 70 % de leur chiffre d'affaires. L'État doit encourager les maires à étendre les terrasses sur le domaine public sans coût supplémentaire. Le tourisme n'est pas qu'une industrie. C'est le miroir dans lequel les Français admirent notre pays et qui fait rêver quelques milliards de personnes à travers le monde. La France brille d'un éclat sans pareil, ne le laissez pas s'éteindre Comme le personnel soignant, les professionnels du tourisme demandent non pas une médaille, mais un soutien sans faille d'un État enfin devenu stratège et protecteur. Êtes-vous prêt, monsieur le secrétaire d'État, à le leur accorder ? La parole est

les communes touristiques sont aujourd'hui les plus fragilisées de toutes nos collectivités. Il convient de prendre en compte cet aspect. En effet, pour relancer l'activité touristique,

Pour que notre saison d'été soit la meilleure possible, de nombreux espaces publics ou privés vont devoir s'adapter, afin de tenir compte de la distanciation sociale. Oui, notre société devra « vivre durablement avec le virus » ! Il est donc urgent de nous y préparer. Au-delà du coût pour les acteurs publics ou privés se pose inéluctablement la question de l'application des procédures et des délais, qui sont, en soi, totalement incompatibles avec la notion d'urgence économique. Dans le respect des règles de l'urbanisme et des principes qui les régissent, les maires seront certainement saisis de demandes qui devront être instruites avec rapidité et avec un sens aigu de l'adaptation.

Par la voie des ordonnances ou de la loi, comme par la voie réglementaire, quelles règles, quels délais envisagez-vous d'adapter ? Quelles prérogatives spécifiques entendez-vous donner aux maires pour en faire les acteurs centraux du redémarrage de notre économie touristique ?

Ses entrepreneurs locaux font vivre nos villages. Leurs établissements sont des points d'attraction souvent indispensables, là où tant de commerces de proximité ont déjà fermé et où le développement économique est le plus fragile. Les mesures prises lors de la phase de confinement et celles annoncées la semaine dernière, que je salue, étaient indispensables. Elles vont indéniablement dans le bon sens, même s'il faudra sans doute encore les ajuster dans les mois qui viennent. Néanmoins, en dépit de ces aides, seule la reprise d'activité permettra d'assurer l'avenir de ces entreprises. L'Italie a passé ce cap hier. En France, il faudra attendre le 2 juin pour les départements classés en vert. Quant à ceux figurant en rouge sur la carte, aucune date n'a encore été arrêtée. Avez-vous davantage d'informations à nous communiquer quant à un calendrier éventuel pour ces En outre, ces femmes et ces hommes courageux, qui ne rechignent pas à la tâche, se préparent, malgré les incertitudes, à accueillir de nouveau des clients dans les meilleures conditions sanitaires possible. Or ce cadre n'a pas encore été défini avec précision. Il doit effectivement permettre d'assurer la sécurité sanitaire des clients sur l'ensemble du territoire national. Cela étant, il doit être souple et retenir des solutions de bon sens, permettant une appréciation au cas par cas par les maires et les préfets afin de tenir compte des réalités locales et de prendre en considération les différentes situations possibles.

On aboutirait à des situations ubuesques : des touristes auraient réservé dans des établissements qui ne pourraient pas ouvrir, du fait de consignes sanitaires trop contraignantes. Enfin, nous n'avons pas de visibilité quant aux moyens. Les mesures concernant le tourisme social se font attendre, alors que la mise en oeuvre rapide d'un soutien aux familles les plus modestes et à tous ceux qui vont faire face à des difficultés nouvelles est absolument nécessaire pour accélérer et renforcer la demande pour cet été. Vous avez aussi annoncé des plans sectoriels. J'appelle votre attention sur le secteur du tourisme fluvial, qui participe à l'économie de nombreux territoires et souffre beaucoup de cette crise. Avez-vous prévu des mesures spécifiques de relance du tourisme fluvial ? Je me félicite de la feuille de route sectorielle annoncée pour le thermalisme ; mais qu'en est-il du report des échéances de crédit, en particulier pour les collectivités territoriales supports d'établissements thermaux ?

le Président de la République a tenu une réunion vendredi dernier afin de préparer les mesures indispensables, qui prendront différentes formes et devraient être annoncées dans la première quinzaine de juin. Je travaille avec les régions

partiellement prises en compte à ce stade. En premier lieu, je pense aux hébergeurs et accueillants individuels. Ils peuvent être labellisés « Gîtes de France », « Clévacances » ou « Bienvenue à la ferme », réseau des chambres d'agriculture. Ils ont beaucoup investi et valorisent un patrimoine naturel et bâti souvent inestimable. Ils assurent un maillage essentiel dans tous les territoires,

Vous comprendrez qu'en tant que sénateur de la Vendée, au même titre que mon collègue Bruno Retailleau, je m'attache au Puy du Fou, que vous connaissez bien, pour bien connaître la Vendée. Deuxième parc français en termes d'affluence, le Puy du Fou est un modèle de développement local reconnu au niveau international. Le Puy du Fou, c'est 2 500 emplois directs, dont 300 permanents en CDI ; c'est 4 500 emplois indirects ; c'est l'accueil, chaque année, de 2,3 millions de visiteurs. Le Puy du Fou, c'est un supplément d'âme qui donne son goût à la France fait rayonner notre histoire au-delà de la Vendée, des Pays de la Loire et du pays tout entier. Le Puy du Fou a proposé un cahier des charges garantissant une ouverture dans des conditions sanitaires irréprochables, pour le personnel comme pour les visiteurs. Ce dossier est sur le bureau du Président de la République, sur celui du Premier ministre et sur le vôtre. Sur ces

Pour autant, elles ne sont pas suffisantes, car le secteur du tourisme et des cafés, hôtels et restaurants est l'un des plus touchés par la crise sanitaire ; or plusieurs secteurs en dépendent. Nous craignons que les mesures de relance annoncées ne profitent qu'aux acteurs les plus solides et les mieux dotés, c'est-à-dire à ceux qui auront encore les moyens d'investir en fin de saison, et aux territoires à forte rentabilité. S'il faut des mesures d'urgence pour assurer le redémarrage, pour reprendre ensuite une pleine activité économique, le secteur aura besoin de lisibilité, de réservations et de revenus, bref, de travail, avant de pouvoir avant de pouvoir faire des projets et d'investir. Pour cela, il faut d'abord des salariés travaillant dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas des saisonniers. Il faut ensuite des clients solvables. Or certains de nos concitoyens ont vu leurs revenus amputés et auront du mal à partir en vacances. Il faut enfin que les territoires dont le tourisme et l'agriculture sont les principales ressources

faut un calendrier de réouverture lisible pour les CHR, et pourquoi pas l'expérimentation d'une ouverture anticipée des cafés-restaurants dans des zones rurales peu denses. Ce sont parfois les seuls commerces dans les petites communes ; leur rôle touristique n'en convient de mettre en oeuvre un véritable statut du saisonnier, qui garantisse une meilleure indemnisation, un suivi social et médical, ainsi que des formations permettant des évolutions de carrière. faut aussi une forte incitation à l'organisation de voyages et de sorties scolaires pendant les prochaines années, et un élargissement exceptionnel des chèques-vacances aux 50 % des Français au-dessous du revenu médian, par un abondement de l'État, ainsi que des collectivités territoriales et des comités d'entreprise apporter un soutien financier aux territoires en zone de revitalisation rurale, dont le tourisme constitue la principale ressource non agricole. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous m'indiquer si le Gouvernement peut, rapidement, mettre en oeuvre ces mesures de relance du secteur du tourisme ?

Les festivals ont payé un lourd tribut à l'épidémie, en étant bien souvent purement et simplement annulés. C'est l'ensemble du monde culturel qui est aujourd'hui plongé dans une profonde angoisse. Même à l'heure du déconfinement, les conditions d'exercice de l'ensemble des activités liées à la saison culturelle estivale demeurent hautement compromises. Une année sans festival priverait nos villes et nos villages d'un lien social fondamental, et c'est une partie de son âme que perdrait notre pays. Il est déjà acté qu'aucune manifestation rassemblant plus de 5 000 personnes ne se tiendra cet été. Pour ces événements, l'unique question est désormais : comment l'État compensera-t-il le colossal manque à gagner Pour les autres, le Gouvernement doit se prononcer le 2 juin, avec la Fête de la musique en ligne de mire. De nombreuses interrogations pèsent encore sur les deux semaines à venir. Au Sénat, dans le cadre du groupe de travail « Création », et sous l'impulsion de notre collègue Sylvie Robert,

Il est parfaitement conscient des enjeux. Les organisateurs souhaitent maintenant des informations précises : il est urgent que l'État fixe un cadre clair, pour la période courant jusqu'à la fin du mois d'août. Quelles règles de protection les structures devront-elles mettre en place pour leurs équipes, qu'elles soient administratives, techniques ou artistiques ? Quelles sont les conditions applicables en matière d'accueil du public ? À ce stade, les annonces du Président de la République ne permettent pas de répondre à ces questions. Le monde de la culture attend des réponses précises et pas des envolées lyriques. Monsieur le secrétaire d'État, l'espoir est immense, la déception le serait aussi.

L'hôtellerie de plein air, c'est 22 millions de visiteurs par an. Je comprends tout à fait la nécessité d'adapter, comme on l'a fait, les autorisations préfectorales aux situations sanitaires locales. Mais je sais aussi que les gestionnaires de campings ont besoin, à très court terme, de clarifications, notamment pour savoir s'ils pourront rouvrir leurs portes dès à présent, pour les ponts de l'Ascension et

des efforts qu'ils devront fournir pour accueillir très prochainement du public. En outre, les mobil-homes loués à l'année sont souvent utilisés comme des résidences secondaires à prix abordable. Accepteriez-vous d'autoriser leur réouverture, au moins pour les locataires domiciliés dans un rayon

aux collectivités qui attendent avec impatience le retour des touristes français, européens et internationaux. Par ailleurs, si je salue les mesures d'accompagnement mises en place au profit des professionnels du secteur touristique, quelques zones d'ombres persistent pour ce qui concerne les voyageurs. Vous avez annoncé un accord européen relatif à la réouverture de l'espace Schengen. Quel est son calendrier et quelle est la position de la France à ce sujet ? Je trouve celle-ci très timide sur ces questions.

je constate que la semaine dernière a plutôt débouché sur des décisions unilatérales. Je pense que cela n'est pas de bonne politique ; il y a vraiment besoin d'évoquer ensemble le rythme de la réouverture des frontières et d'éviter que les uns

Comme l'a souligné notre collègue Michel Raison, la plupart des dispositions prises par le Gouvernement rejoignent les recommandations formulées par la cellule de veille et de contrôle de la commission des affaires économiques du Sénat, qui a procédé à des dizaines d'auditions et recueilli les retours de nombreuses entreprises de proximité sur tout le territoire

filière touristique à part entière, qui cumule les difficultés liées au manque de main-d'oeuvre et à l'absence de touristes. Je demande au Gouvernement d'intervenir pour étendre, à cette filière, les dispositifs d'aides d'urgence. Vous le voyez, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à l'issue de notre débat, de nombreux points restent encore à éclaircir. Les difficultés du secteur des transports ont été évoquées, avec, notamment, la question du remboursement des vols annulés. qui a choisi d'autoriser la pratique des avoirs pour protéger la trésorerie des compagnies aériennes, est en infraction avec la réglementation communautaire. Je compte donc sur le Gouvernement pour obtenir

les professionnels ont d'ores et déjà besoin de dates, pour constituer des stocks, recruter des saisonniers et assimiler les normes qu'ils devront respecter. Chaque jour qui passe se traduit par des pertes énormes. Ainsi, les cafés et restaurants, qui attendent l'autorisation de reprendre leur activité, s'inquiètent à juste titre des mesures envisagées par le Gouvernement.

Prendre les transports en commun me semble autrement périlleux ; pourtant, c'est le quotidien de nombreux Français, qu'ils soient en zone verte ou en zone rouge. Sur tous ces sujets, nous avons besoin de bon sens, de clarté. on peut regretter le flou ayant entouré la réouverture de certains lieux culturels. Depuis le 11 mai dernier, les « petits » musées et les « petits » monuments ont pu rouvrir ; les grands restent fermés. Cette distinction vague me semble peu justifiée, dès lors que de grands musées, tels ceux de la capitale, envisagent de mettre en oeuvre des dispositifs drastiques de protection des visiteurs. Certaines expositions sont annulées, faute de connaître la date où elles pourraient être reportées. De même, les théâtres et les cabarets ne peuvent mettre en place leur saison, ce qui affecte l'ensemble d'une filière déjà éprouvée par les grèves contre la réforme des retraites. Autre incohérence, signalée pendant ce débat : à l'inverse des parcs animaliers et des aquariums, dont la réouverture est possible, même en zone rouge, sur décision du préfet, les parcs d'attractions n'ont aucun horizon. La plupart de ceux-ci travaillent pourtant en plein air et ont déjà prévu un protocole sanitaire

il y a urgence, et les prochaines semaines seront décisives. Lors de ce débat, nous avons tous, dans cet hémicycle, voulu montrer combien l'ensemble du territoire est concerné. Par sa géographie, son patrimoine et ses savoir-faire, notre pays, la France, est la première destination mondiale pour le tourisme. Aujourd'hui, ce que nous devons défendre, c'est cet art de vivre que le monde nous envie, l'ADN français.

et de la communication, portant sur les modalités de réouverture des établissements d'enseignement ainsi que sur les conditions d'organisation des concours et examens et de préparation de la prochaine rentrée scolaire.

la mise en place de l'école à distance. Nous avons également eu des discussions sur l'élaboration de la carte scolaire ; sur ce sujet, vous avez d'ailleurs écouté le Sénat, et je vous en remercie. Tout cela, c'était trois jours avant l'annonce, par le Président de la République, de la réouverture des établissements scolaires à compter du 11 mai, nous prenant tous un peu de court, je dois le à commencer par les premiers partenaires de l'éducation nationale, les collectivités territoriales, que nous représentons ici. Quelles que soient leurs interrogations, ces dernières restent formidablement engagées

se sont organisés en un temps record pour offrir aux enseignants et aux enfants les conditions de la reprise. À cet égard, nous sommes heureux d'avoir pu régler la question de leur responsabilité particulière ainsi que celle des directeurs d'école, lors des débats sur la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire nous ne saurions trop insister : une reprise réussie pour notre école et nos enfants nécessite une vraie concertation. Le couple maire-préfet, plus largement les élus locaux et les représentants de l'État doivent travailler ensemble. Ils l'ont fait ces derniers jours, j'ai pu le constater dans le département dont je suis élue, où 90 % des écoles rouvrent progressivement et à leur rythme. De l'avis même des élus, cela se passe plutôt bien avec les instances académiques, même là où les maires ont choisi de ne pas rouvrir.

Je suis heureuse de la tenue de ce débat, et je remercie la conférence des présidents du Sénat d'avoir accepté de l'inscrire à l'ordre du jour en plein coeur de l'actualité. Cela nous permettra d'échanger, de remonter remarques et inquiétudes et d'avoir vos réponses. Pour conclure, je veux saluer

la commission de la culture a mis en place un groupe de travail sur l'enseignement scolaire, que j'ai eu l'honneur de piloter. Je remercie notre présidente et le bureau de notre commission de cette initiative, et je salue l'ambiance de travail, excellente bien que studieuse, de notre groupe transpartisan mais néanmoins intéressant. Nous avons élaboré onze préconisations, qui ont fait consensus parmi les différents groupes politiques. Celles-ci s'articulent autour de cinq idées principales : méthodologie, concertation, souplesse, adaptation aux réalités des territoires et préparation de la prochaine rentrée, en tenant compte des circonstances exceptionnelles qui ont marqué l'année 2019-2020. La crise sanitaire que nous traversons et les mesures prises pour y faire face sont, de mémoire d'hommes, inédites en France et chez nos principaux partenaires. Certes, les écoles ont dû fermer pendant de longues semaines à Saint-Martin, à la suite du passage de l'ouragan Irma, mais jamais, au grand jamais, l'intégralité des établissements scolaires n'avait fermé de manière inopinée, sur l'ensemble du territoire, pour une période aussi longue, même pendant la pandémie de la grippe espagnole survenue il y a cent ans, occasionnant 250 000 morts près de 50 millions de décès dans le monde. Pendant les deux guerres mondiales, il n'y a pas non plus eu d'injonction de fermeture généralisée des établissements scolaires. L'obligation d'instruire prévalait ; c'est un régulateur social. C'est dire la situation particulière à laquelle a dû faire face le personnel de l'éducation nationale, le vendredi 13 mars dernier. Je salue d'ailleurs l'extraordinaire mobilisation et l'adaptation dont ont fait preuve le ministère de l'éducation nationale, vous-même, monsieur le ministre, et des enseignants pour répondre au plus vite à cette crise et permettre une continuité pédagogique pour la grande majorité des élèves.

Elle ne s'est pas faite sans questionnements, sans incertitudes et, parfois, sans certaines tensions, avec les élus locaux, les familles et les autorités déconcentrées de l'État- préfet et éducation nationale. Je ne reviendrai pas sur la notion de responsabilité des maires.

à la concertation et à une écoute réciproque. Sous certains aspects, cette crise a permis d'améliorer les liens entre ces différents acteurs. Certes, cela reste perfectible, mais on constate des progrès. De manière générale, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dresser un premier bilan de la réouverture des écoles primaires ? Combien d'écoles ont rouvert et, surtout, quel est le pourcentage d'élèves du primaire accueillis ? Quelles sont les perspectives pour les collèges qui sont en train de rouvrir dans les départements classés en zone verte ? Je tiens à vous signaler plusieurs difficultés partagées par de nombreux directeurs d'école : comment choisir les élèves à accueillir prioritairement ? Une circulaire sur ce sujet est-elle prévue ? Par ailleurs, certains enseignants ou Atsem ne peuvent pas retourner travailler, en l'absence d'un accueil par l'école de leurs enfants. Il nous faut des directives et une organisation nationale, comme le disait le maire de Pontarlier. J'en viens à l'objectif de cette réouverture des classes, non pour les élèves- ce point sera très certainement abordé par mes collègues dans le cadre de leurs nombreuses questions -, mais pour l'institution scolaire. La reprise très progressive, échelonnée, des cours doit permettre de tirer des enseignements pour l'organisation des cours dans les semaines à venir, mais aussi pour la rentrée de septembre 2020. En effet, même si la recherche fait chaque jour d'énormes progrès en matière de connaissance de ce virus, il n'y a pas de perspective de vaccin ni de traitement à si court terme, et nous sommes encore très loin de l'immunité collective. Quelles sont donc les pistes de réflexion de votre ministère pour la rentrée scolaire de 2020, dans l'hypothèse où le virus serait encore en circulation sur le territoire, même avec un R0 très faible ?

Serait-il envisageable de mettre en place un enseignement mixte entre présentiel et enseignement à distance, notamment pour les classes les plus grandes, les lycéens par exemple, voire pour les collégiens et les primaires ? Ce système pourrait s'appuyer sur une brigade d'enseignants dédiés

Un tel système nécessiterait toutefois un important travail de concertation avec l'équipe pédagogique en présentiel et une mutualisation à l'échelle du territoire. Il implique en outre un équipement et une infrastructure informatique performants et disponibles pour les enseignants et les élèves, afin de ne pas accentuer les inégalités. Des réflexions sont en cours avec les collectivités locales et les principaux opérateurs de la téléphonie et du numérique, pour lutter contre la fracture numérique. Cela fera l'objet d'une question de mon collègue Stéphane Piednoir.

prospective que vous venez de suggérer, puisque nous devons avoir une approche cohérente de tout ce qui s'est passé. Pour ma part, je raisonne en quatre temps. La première période a été le confinement, commencé le 15 mars dernier et achevé le 11 mai.

puis pour l'Oise, pour le Morbihan, pour le Haut-Rhin et puis pour la France entière. On a parfois commenté mes propos quand j'ai indiqué, après l'annonce du Président de la République du 12 mars : « nous sommes prêts ».

au fil du temps les choses. Madame la présidente de la commission, vous avez rendu hommage aux professeurs, mais aussi à l'administration, et je vous en remercie. Il est toujours facile d'attaquer l'administration de l'éducation nationale-

au milieu des difficultés très particulières que nous rencontrions. Je le souligne, parce que l'on a parfois l'impression que les choses se déroulent tout naturellement, comme par magie. Non, il y a tout simplement du personnel administratif, parfois un peu

toutes nos forces et toutes nos faiblesses sur le plan technologique, qui nous permettront de nous améliorer dans le futur. Le déconfinement- la période dans laquelle nous sommes actuellement -est aussi un moment tout à fait exclusif, inédit. Jamais l'éducation nationale, dans toute son histoire, n'a eu à faire ce que nous sommes en train de faire, non une rentrée, mais ce que nous avons préféré appeler « une reprise

découverte, pour que les enfants reviennent à l'école. Il y a déjà suffisamment de dégâts sociaux liés au confinement pour ne pas en ajouter en attendant davantage. Une autre perspective serait l'école « garderie », un moment où l'on s'occupe juste de garder les enfants. Je suis farouchement opposé à cette approche également. Les deux approches- rien du tout ou l'école garderie -sont délétères pour l'idée qu'on peut se faire de l'école de la République. Il faut que les enfants soient là pour apprendre, même si c'est dans des circonstances particulières.

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

Prendre cette décision fut difficile, car il s'agit d'un fondement notre République. Nous commençons à les rouvrir. Nous savons combien cet exercice est complexe, complexe, monsieur le ministre, pour vous et surtout pour les maires, pour les directeurs et directrices d'école et pour les professeurs. Cette situation inédite nous a contraints à mettre entre parenthèses le respect d'un principe important de notre école républicaine : l'obligation. Alors que nous débattons des modalités de réouverture des établissements, je souhaite redire ces mots de Jules Ferry sur l'inscription dans la loi de l'obligation scolaire : « Nous mènerons à bien cette grande réforme, qui est à la fois la plus grande des réformes sociales et [ ...] la plus durable des réformes politiques ... Lorsque toute la jeunesse française se sera développée, aura grandi, triple étoile de la gratuité, de l'obligation et de la laïcité, nous n'aurons plus rien à craindre des retours du passé. » Si nous pouvons comprendre pourquoi il a fallu suspendre l'obligation scolaire, nous conviendrons toutes et tous qu'il est urgent de trouver comment réunir les conditions pour que nous puissions la rétablir au plus vite. C'est nécessaire pour ne pas accroître les inégalités entre les familles, et surtout pour réussir à accompagner les décrocheurs scolaires efficacement. Je crois que nous en serons capables collectivement. Notre groupe de travail « enseignement scolaire » l'a prouvé en fournissant un travail transpartisan et constructif. Pour la fin de cette année scolaire, l'enjeu est de pouvoir accueillir chaque enfant. C'est impossible dans nos seuls locaux scolaires. Il faudra donc s'appuyer sur nos collectivités locales, mais il est impensable de leur demander cela sans leur donner les moyens adéquats. Monsieur le ministre, je souhaite que vous précisiez comment les collectivités locales vont être accompagnées financièrement

et du décrochage scolaire. C'est indispensable pour réaliser les aménagements pédagogiques nécessaires et trouver des solutions pratiques adaptées à chaque contexte. Pouvez-vous nous indiquer si ce bilan complet est prévu ? La parole est à M. le ministre. Madame la sénatrice,

qu'une contrainte forte, une circonstance négative, peut amener des évolutions positives si nous travaillons bien. Nous avions de toute façon pour objectif de développer, en lien avec les collectivités, la place du sport et de la culture à l'école. Le dispositif 2S2C,

et l'ensemble des sénateurs du groupe RDSE. Depuis le 11 mai, les écoles rouvrent progressivement dans notre pays. Ce retour à l'école des élèves s'organise selon un protocole sanitaire exigeant, lourd et complexe. Or, pour mettre en place ces mesures absolument nécessaires, les communes ne sont pas égales en termes de moyens

Les communes font au mieux avec les ressources dont elles disposent, mais les mesures sanitaires entraînent de lourdes dépenses qui vont durement peser sur les finances des municipalités, d'autant que la situation actuelle risque de perdurer jusqu'à la rentrée de septembre. Alors que les nouvelles équipes municipales élues au premier tour vont entrer en fonction, les élus des petites communes ont besoin d'être soutenus. Monsieur le ministre, comment comptez-vous aider concrètement les petites communes et les communes en situation financière difficile à

La réouverture des écoles et la rentrée scolaire sont des enjeux cruciaux du déconfinement au regard de la continuité éducative pour nos enfants. Vendredi 8 mai, vous avez indiqué, monsieur le ministre, que la formule de classes par demi-groupes pourrait être reconduite en septembre et que l'enseignement à distance continuerait à jouer un rôle très important. Il s'agit en effet de concilier deux exigences : la réussite éducative de nos enfants et la protection sanitaire, au moment où une crise sans précédent frappe notre pays. Je souhaite attirer votre attention sur une problématique majeure à laquelle nous sommes confrontés : celle de la fracture numérique au sein de notre système éducatif et des inégalités scolaires qu'elle engendre. Connexion internet défaillante, familles dépourvues d'ordinateur et d'imprimante : dans les zones rurales comme dans les quartiers populaires, les élèves sont parfois dans l'impossibilité de suivre les enseignements dans de bonnes conditions. Malgré le travail considérable des associations et la mobilisation des enseignants et des pouvoirs publics, cette fracture engendre de lourdes conséquences sur la réussite éducative de nos enfants.

quelles mesures mettrez-vous en place à la rentrée scolaire pour renforcer la continuité éducative et lutter contre le décrochage scolaire ? La parole est à M. le ministre.

La réouverture des établissements, depuis le 11 mai, s'est faite selon le même style hasardeux : l'impréparation pour la sortie de confinement a fait suite à l'impréparation pour l'entrée en confinement, sans aucune concertation avec les collectivités locales. Il eût été plus pertinent et plus efficace

La situation dans ma ville est d'autant plus critique que les élèves, à Marseille, ne craignent pas seulement le virus : ils ont surtout peur que le plafond leur tombe sur la tête, qu'il n'y ait pas d'eau courante, que la chaleur les étouffe en été ou que le froid les fasse grelotter

Puisque vous avez choisi de vous défausser sur les maires, une trentaine d'entre eux sur cent dix-neuf, dans mon département, ont décidé de ne pas rouvrir les écoles. Ils ont peur pour les enfants, pour le personnel, pour les parents, mais aussi pour eux-mêmes, car c'est le maire qui sera tenu pour responsable si un seul enfant, enseignant ou agent municipal est contaminé Vous avez menti à tous les Français, et maintenant vous vous cachez derrière les maires de France. C'est simple : le jour où l'on n'aura besoin de rien, on saura que l'on peut compter sur vous ! En attendant, les Français et leurs maires, le pays réel,

et qu'ils pourront retrouver une place centrale dans l'organisation de la vie de la Nation ?

par des protocoles sanitaires extrêmement complexes, élaborés tardivement et auxquels les collectivités territoriales ont dû se plier très rapidement, ne remédie pas aux inégalités sociales. Dans mon département de la Seine-Maritime, par exemple,

de la mi-juin à la fin juillet et les concours internes à la rentrée, de manière à préserver les droits de ceux qui les ont préparés. La parole est à Mme Colette Mélot.

ainsi que par les partenaires de celle-ci que sont les collectivités, dans cette situation tout à fait inédite. Le Gouvernement a annoncé qu'une priorité serait accordée à l'accueil des enfants porteurs d'un handicap par les établissements scolaires. En effet, les enfants atteints de troubles cognitifs et leurs familles ont particulièrement souffert des effets du confinement- rupture de soins, perte de repères liée aux changements d'habitude, épuisement des familles si bien que le retour à l'école était très attendu des parents comme des enfants. Pourtant, en dépit des annonces du Gouvernement, on a pu constater, dans un certain nombre d'écoles, que des parents d'enfant porteur d'un handicap se heurtaient à un refus d'admission. Les exemples ne manquent malheureusement pas. La raison principale invoquée serait l'impossibilité, pour ces enfants, de respecter les gestes barrières. Les associations de défense des personnes handicapées et les fédérations de parents d'élèves plaident pour que le Gouvernement garantisse un droit à l'éducation pour tous les enfants. Il est regrettable de devoir constater que les enfants les plus fragiles sont les premières victimes du déconfinement.

Pour autant, le protocole sanitaire souligne qu'une attention particulière doit être apportée aux personnes en situation de handicap ou porteuses de maladies évoluant sur une longue période. alors que le Gouvernement affiche clairement sa volonté de bâtir une école inclusive, conformément au souhait des parents d'élèves et des fédérations d'associations de défense des personnes en situation de handicap, êtes-vous prêt à mettre en oeuvre des mesures concrètes permettant d'accueillir ces enfants dans de bonnes conditions ?

Lors de la présentation des modalités de sortie du confinement, le Premier ministre a bien mentionné que la réouverture des lycées était conditionnée à la situation sanitaire mais que, en tout état de cause, elle n'interviendrait pas avant le début du mois de juin,

Nous avons bien compris que vous aviez le souci de maintenir un certain climat de stimulation pour les élèves, afin que la période actuelle ne soit pas inutile. Toutefois, je crois qu'il est temps de dire

se sont désengagés de leur scolarité depuis le début du confinement. Il ne s'agit pas des élèves dont l'institution scolaire n'a aucune nouvelle- les 4 % de décrocheurs -, mais d'élèves ne communiquant que faiblement avec leurs professeurs. Cette proportion atteindrait 30 % dans les collèges en REP et les lycées professionnels. le confinement a une incidence importante sur l'acquisition et la consolidation des apprentissages. Conscient de ce problème, votre ministère s'est déjà fortement engagé. Je pense notamment au soutien scolaire à distance mis en place pendant les vacances de printemps. Votre circulaire du 4 mai dernier semble dessiner trois temps : la période de la reprise des cours, jusqu'au 4 juillet ; les vacances d'été ; la rentrée de septembre prochain. Ma question porte sur les deux dernières périodes.

en fonction des classes ou des difficultés scolaires ? En ce qui concerne la rentrée de 2020, la circulaire indique que l'année scolaire 2020-2021 devra ménager, jusqu'aux vacances de la Toussaint, des temps pour consolider les apprentissages. Peut-on aller plus loin et prévoir une adaptation des programmes et un lissage par cycle ? Enfin, la circulaire de rentrée 2019 avait été publiée le 28 mai 2019. Pouvez-vous nous donner une échéance indicative pour la publication de la circulaire de rentrée 2020 ? Est-ce une question de jours, de semaines ? Sera-t-elle publiée avant le début des vacances d'été ? La parole est à M. le ministre. Monsieur le

C'est pour ces enfants-là que vous rouvrez les écoles, mais ce sont ceux-là qui ne sont pas revenus ... Ainsi, dans mon village, certains parents ne se sont même pas donné la peine de répondre aux professeurs sur leur souhait de remettre ou non leur enfant à l'école le 14 mai ; bien sûr, ils n'étaient pas présents à la rentrée, jeudi dernier-

ou plutôt toucher leurs parents ? Les services sociaux sont un premier relai, mais nous savons qu'il est insuffisant, surtout s'il s'agit d'inscrire ces enfants pour l'été 2020.

chacun de nous a pu mesurer, dans son département, la profonde et légitime inquiétude des maires devant le poids des responsabilités qui pèsent sur eux. Complexe, elle l'est également pour les responsables éducatifs et les enseignants, compte tenu de la nécessité pour eux de réorganiser totalement l'accueil des élèves et les activités scolaires. l'est enfin pour les parents, tiraillés entre le désir de protéger leurs enfants et celui de retrouver une activité professionnelle aussi normale que possible. Dans ce contexte, qui nous oblige à la rigueur des procédures et à la protection de tous à l'égard du virus, la situation des enfants handicapés est quelque peu passée à l'arrière-plan. Une fois encore, ce sont les plus fragiles que l'on oublie trop facilement lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ... Je voudrais évoquer, sans pathos mais avec réalisme, la situation vécue par Liam, un jeune autiste de 11 ans scolarisé en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) à Morsang-sur-Orge, dans mon département, et que je suis depuis plusieurs années. Deux mois de confinement auront suffi à lui faire perdre tous ses repères, son environnement matériel et affectif, ainsi que les progrès accomplis au prix de tant d'efforts. Liam présente aujourd'hui des signes de régression et est devenu agressif.

peut avoir des effets extrêmement négatifs pour les élèves en situation de handicap. Le cas de l'autisme est très significatif à cet égard. C'est l'une des raisons pour lesquelles

est à Mme Claudine Lepage. Monsieur le ministre, les établissements d'enseignement français à l'étranger sont durement touchés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19.

non titulaires de l'AEFE, dans la mesure où leur année de stage doit être effectuée en France. Dans quelles conditions seront-ils affectés et pourront-ils s'installer en cours d'année ? Par ailleurs, du fait de la fermeture des frontières, des contingences aériennes et des quatorzaines mises en place à l'arrivée, les candidats admissibles en poste à l'étranger ne sont pas certains de pouvoir se présenter aux épreuves d'admission en septembre. Pourquoi le ministère n'applique-t-il pas aux concours internes les mesures exceptionnelles qu'il a prises pour les concours externes, soit l'admission sur la base des épreuves d'admissibilité ?

Vous avez mentionné le taux de 5 % de décrocheurs au cours des deux derniers mois. Ce chiffre paraît pour le moins sous-estimé, quand on sait que 1,8 million d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté en France.

Monsieur le ministre, depuis la rentrée du déconfinement, les enseignants des quartiers populaires nous alertent : les victimes collatérales du confinement, à savoir les décrocheurs scolaires, ne reviennent pas

Des villes l'ont déjà entreprise, en s'appuyant sur les centres sociaux ou des associations. Monsieur le ministre, comment comptez-vous répondre à cette situation sur les plans pédagogique, psychologique et social ? L'année scolaire 2020-2021 ne peut pas être préparée de la même façon les autres. Êtes-vous prêt à lancer avec toute la communauté éducative, les associations et les collectivités territoriales concernées- régions, départements, villes -une grande concertation déconcentrée pour élaborer une réponse à la hauteur de l'enjeu qui est devant nous,

sachant que la rentrée du 11 mai reposait sur trois piliers totalement inédits : le volontariat parental, la mise en place dans tous les bâtiments accueillant les écoliers d'un protocole plus que draconien

rentrée il y eut, ce fut à effectifs très restreints, des parents inquiets préférant que leurs enfants restent à la maison. Cette reprise s'est-elle bien passée ? Pas toujours, notamment pour les plus petits, pour qui le retour à l'école s'est transformé en un nouveau confinement, dans leur classe. Aussi une question revient-elle inlassablement chez les élus, mais aussi chez de très nombreux parents et enseignants

La crise sanitaire que traverse le pays a conduit le Gouvernement à reporter les examens nationaux et les concours. Concernant les trois filières de classes préparatoires aux grandes écoles, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal, a annoncé, le 17 avril dernier, que les écrits des concours seraient reprogrammés entre le 20 juin et le 7 août prochain. La question des conditions et des lieux de leur organisation doit donc être résolue. Il s'agit notamment de préparer les centres d'examen ou lycées habituels pour accueillir les étudiants à ces dates, en s'assurant que les consignes sanitaires seront bien respectées, pour ne pas mettre les candidats ni les surveillants en danger. Dans cette optique, le service des concours des écoles d'ingénieurs essaie d'ouvrir davantage de centres, afin de limiter les déplacements pour les étudiants. Au lieu d'ouvrir des centres, il a été envisagé, dans certaines académies, que les étudiants passent les épreuves de leur concours à Paris. On voit que, sur le terrain, la gestion du nouveau calendrier soulève d'importantes difficultés. N'aurait-il pas fallu vérifier que ce calendrier est concrètement tenable avant de l'imposer sur nos territoires et à nos lycées ?

ce point par notre commission, le ministre de la culture avait renvoyé aux collectivités territoriales. Cela ne suffit pas. Je rappelle que l'État dispose de la compétence pour les cursus,

en partenariat avec les collectivités locales et les fédérations d'éducation populaire, à la mise en place de ces colonies de vacances et séjours de loisirs. Bien évidemment, de nombreuses questions demeurent, tenant à l'évolution de l'épidémie et des traitements, ainsi qu'aux modalités d'organisation et aux moyens humains et financiers pour les collectivités territoriales. Cette crise sanitaire a également entraîné une accélération considérable de l'entrée du numérique dans la pédagogie. L'éducation L'éducation nationale s'est adaptée à marche forcée, les enseignants essayant de trouver des solutions pour garder le contact avec leurs élèves et continuer à faire cours, en se formant parfois

pour permettre aux enseignants de compléter et d'actualiser leurs connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques ». C'est dans cet esprit que, avec Max Brisson, nous avions renforcé le volet numérique de la loi pour une école de la confiance. Cette période a également été l'occasion, monsieur le ministre, d'innovations pédagogiques, de mise en place de nouvelles façons de travailler, de modifications

et à développer. Toutefois, sans accompagnement ni réflexion, l'intégration du numérique à l'école risque, malgré elle, de creuser les inégalités entre élèves, entre professeurs et entre territoires. L'apprentissage à distance mis en place depuis le 16 mars

notre séance se déroule dans les conditions de respect des règles sanitaires mises en place depuis le mois de mars. L'hémicycle fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection avant et après chaque séance. Les micros seront désinfectés après chaque intervention. J'invite chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité. Je rappelle également que les sorties de la salle des séances devront exclusivement s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle. Je rappelle que tous les orateurs, y compris le Gouvernement, s'exprimeront depuis leur place, sans monter à la tribune. Je rappelle, enfin, que, afin de limiter la circulation de documents, vous êtes invités à utiliser vos tablettes et la fonctionnalité « En séance sur notre site internet pour prendre connaissance du dérouleur et des amendements. Des liasses resteront à votre disposition sur demande. Dans la discussion générale, la parole est à M. Bruno Retailleau, auteur

que les frais qu'elles doivent engager soient insuffisamment couverts par le régime de sécurité sociale ? Est-il juste que l'on durcisse les conditions de prise en charge des soins

qui donnent de leur temps pour leurs compatriotes au sein des conseils consulaires ou de l'Assemblée des Français de l'étranger ne disposent pas des moyens, du soutien, de l'accompagnement et, pour tout dire, de la reconnaissance dont bénéficient les autres élus en France ? Non, mes chers collègues, rien de tout cela n'est juste

sans exception et sans considération de leur choix de lieu de vie, la même protection et la même attention. C'est au nom de cette attention que nous leur devons que notre groupe

mais également de revenir à un taux minimum d'imposition de 20 %, contractuellement de 30 %, sur les revenus de source française lorsqu'ils dépassent la limite supérieure de la deuxième tranche.

de leur situation par rapport à leur patrie ? Il leur est recommandé de rester dans leur pays d'accueil. Ainsi, les expatriés ne sont plus chez eux nulle part ; ce sont des étrangers partout. Les Français établis hors de France ne bénéficient évidemment pas des lois françaises en matière de chômage partiel, d'aides sociales ou d'aides aux entreprises. Le plan de 240 millions d'euros annoncé par le Gouvernement est utile, mais très insuffisant pour faire face à la crise. Les Français résidant hors de France participent au rayonnement international de notre pays sur les plans économique, culturel ou linguistique. Loin des stéréotypes, ce sont de petits retraités, de jeunes entrepreneurs, des créateurs de start-up, des salariés d'entreprises françaises ou locales ou encore des médecins, des chercheurs, des étudiants Malheureusement, ils sont depuis des années considérés comme des citoyens de seconde zone. Il y a les Français qui résident dans l'Hexagone et dans les outre-mer, qui eux sont des Français à part entière, et il y a les Français résidant hors de France. Là encore, il y a deux catégories : ceux qui résident au sein de l'Union européenne et les autres, qui ne sont pas traités de la même manière. Comme nos budgets sont toujours contraints, les premiers touchés par les réductions de crédits sont les Français de l'étranger. face à ces difficultés, nous proposons un plan d'action qui recouvre cinq grands thèmes : le régime fiscal, le réseau diplomatique, la représentation politique, le réseau éducatif et la protection sociale. premier sujet, nos objectifs sont clairs. Il s'agit de revenir sur des décisions injustes et confiscatoires que le Gouvernement a prises en 2019 et qui sont synonymes de régression pour nos compatriotes

Je commencerai par la réforme de l'impôt sur le revenu de 2019. Le Gouvernement a fait voter l'augmentation du taux minimum d'imposition sans clause libératoire. Les revenus sont donc imposables dès le premier euro. Plusieurs compatriotes m'ont indiqué que, avec cette réforme, leur imposition augmenterait de plus de 200 % ... Qui accepterait une telle situation en France ? Un moratoire partiel d'un an a dû être décidé.

Avec le cumul des mesures fiscales et sociales récentes, il pourra se voir prélever plus de 45 % sur ses revenus de source française ; sa pension de retraite sera donc quasiment divisée par deux.

l'aide sociale. Il aura fallu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne pour que le Gouvernement finisse par supprimer, sous la contrainte, la CSG et la CRDS pour les Français résidant dans un État membre de l'Union européenne.

les autres, qui continuent à payer les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine alors qu'ils ne bénéficient d'aucune prestation sociale. Nous proposons donc d'exonérer l'ensemble des non-résidents de CSG et de CRDS sur leurs revenus de source française.

atteint ... De même, les expatriés ne bénéficient pas de la suppression de la taxe d'habitation. Leur domicile en France est assimilé à une résidence secondaire. Ils sont pourtant susceptibles de devoir rentrer rapidement chez eux en France, en particulier en période de crise sanitaire ou politique, ou en cas de perte d'emploi ou de catastrophe naturelle. Concernant l'évolution des services rendus par les ambassades et les consulats, nous bénéficions d'un réseau consulaire de grande qualité, servi par des fonctionnaires dévoués, que je remercie très chaleureusement : malgré la diminution constante de leurs moyens et une augmentation du nombre de Français résidant à l'étranger, ils parviennent, au prix d'un grand dévouement, à assurer un service que l'on peut qualifier d'excellent.

Le ministère de la justice s'est toujours refusé à autoriser les Français de l'étranger à signer des actes notariés par visioconférence, au prétexte d'une trop grande complexité et d'un manque de sécurité.

Nous comptons donc sur le ministère de la justice pour en pérenniser la mise en oeuvre le plus rapidement possible. Nous rencontrons aussi d'énormes difficultés s'agissant de la légalisation des certificats de vie que les retraités établis hors de France doivent fournir chaque année à leur caisse de retraite.

Depuis quelques mois, les directives données à nos postes diplomatiques imposent que ces certificats soient authentifiés non plus par eux, mais par les autorités locales, ce qui ajoute de la complexité. Nous proposons que les certificats de vie puissent à nouveau être visés par nos postes diplomatiques et par les mairies françaises.

Pendant des périodes difficiles comme celle que nous vivons, nous pouvons constater à quel point le rôle des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires est capital. Ils sont nos yeux et nos oreilles sur place. Ils nous alertent sur les situations souvent dramatiques vécues par nos compatriotes. Le texte de la commission conforte les conditions d'exercice de leur mandat, en particulier la prise en charge des frais de transport, la validation des acquis de l'expérience et la reconnaissance officielle de leur mission dans l'ordre protocolaire des postes. L'organisation des élections consulaires, initialement prévue au mois de mai dernier, constitue donc un enjeu essentiel. Nous attendons des réponses du Gouvernement sur ce point. En matière d'éducation, il est proposé de créer des bourses spécifiques pour l'accueil des enfants en situation de handicap lorsqu'ils n'ont pas pu être pris en charge dans le réseau français.

En 2018, l'imposition des 223 674 foyers fiscaux non résidents a représenté 1,3 milliard d'euros, ce qui n'est pas négligeable. tel défaut d'information est source d'idées reçues sur les Français expatriés : on confond bien souvent les de Londres avec les serveurs de Temple Bar Bar ! D'autre part, j'ai pu me rendre compte que la fiscalité applicable aux non-résidents était excessivement complexe. Je l'ai qualifiée en commission de « demi-maquis fiscal » ; nous avons délocalisé notre meilleure usine : l'usine à gaz fiscale gaz fiscale ! Or la simplification du quotidien fiscal de nos compatriotes expatriés ne passe pas uniquement par des modifications législatives. Nous pourrions en effet réfléchir à la mise en place d'un guichet unique et à une clarification de l'application des conventions fiscales.

permet, je le crois, de faire face à ce stade aux conséquences de la crise économique qui suit la crise épidémique. Le troisième sujet, qui n'est pas le moindre, concerne l'école.

Même si la probabilité de l'inscription de ces dispositions dans la loi est mince, nous sommes déterminés à profiter de cette occasion pour évoquer en séance un certain nombre de sujets sensibles pour les Français vivant hors de France, en ce moment de crise très aiguë et particulièrement grave pour eux.

La crise sanitaire actuelle est mondiale. Elle touche les 3 millions de Français installés à l'étranger, souvent dans des pays qui ne connaissent pas nos amortisseurs sociaux. Une perte de revenus, une perte d'emploi, et c'est parfois la perte de l'assurance maladie, voire du droit au séjour. Vous avez annoncé des dispositifs d'accompagnement, mais leur mise en oeuvre laisse dubitatif. Faut-il attendre d'être à la rue, au sens littéral du terme, pour pouvoir faire appel aux services sociaux des consulats ?

Les Français vivant à l'étranger constituent la trame de notre réseau d'influence et de notre présence à l'international. Alors que tout le monde parle de souveraineté, rappelons qu'il n'y a pas de réelle souveraineté sans rayonnement à l'international. Il faut donc préserver nos réseaux et soutenir ceux qui les animent : nos Alliances françaises, les chambres de commerce, les entreprises créées par des Français, vectrices d'emplois en France et aujourd'hui fragilisées. Nous avons formulé de nombreuses propositions sur ces sujets. Que fait le Gouvernement à cet égard ? concerne les bourses scolaires et l'AEFE, des annonces ont été faites. Nous restons dubitatifs quant à la démarche relative à l'Agence, car il ne s'agit que d'une autorisation d'endettement de celle-ci, si l'on se réfère aux documents proposés au conseil d'administration de l'AEFE. Il faudra en effet que les établissements scolaires, donc les familles, remboursent les avances consenties aujourd'hui. Enfin, même si nous avons connaissance des annonces, nous ne sommes pas directement destinataires des décisions finales. Nous les apprenons « par la bande », et elles sont appliquées de manière très hétérogène par les postes. Du fait de notre rôle de contrôle de l'action du Gouvernement, mais aussi parce que les conseillers consulaires ont besoin de ces informations pour remplir correctement leur mission, nous souhaitons obtenir directement ces informations. En cet instant, je veux saluer le travail de nos consulats à l'étranger en matière de rapatriement des Français, en

à l'expatriation, participent au rayonnement et à la renommée de la France à l'étranger. Partout dans le monde, ils sont l'image de notre pays, en particulier de sa culture, de sa langue et de son savoir-faire économique. Aussi, nous devons nous employer, d'une part, à faciliter le quotidien des Français de l'étranger, et, d'autre part, à assurer le maintien de leur lien civique avec l'Hexagone. Cette nécessité d'accompagner nos concitoyens de l'étranger dans leurs démarches nous apparaît encore plus impérieuse à la lumière de la crise épidémique. La fermeture des frontières et des établissements scolaires a posé des difficultés à certains d'entre eux. Les ambassades se sont mobilisées autant qu'elles le pouvaient pour faire face, dans un contexte inédit. Cet épisode me conduit à rappeler l'importance de maintenir un réseau diplomatique dense, disposant des moyens à la hauteur des missions qu'on lui assigne. Comme vous le savez, mes chers collègues, dans le cadre du programme Action publique 2022, le réseau de l'État à l'étranger se réforme, avec une trajectoire de réduction de sa masse salariale. Si un objectif de rationalisation peut être fixé pour nos services publics à l'étranger, il faut que ceux-ci soient toujours en mesure de faire preuve de réactivité en cas de crise. En attendant, la proposition de loi s'attelle- avec une certaine ambition, il faut le dire -à permettre aux Français expatriés de « vivre mieux », selon les mots de son auteur. Mon groupe souscrit bien entendu à ce principe, pour les raisons que je viens d'évoquer. Une partie du texte vise à améliorer la représentation démocratique des Français établis hors de France. Cela a été dit, les dispositions proposées s'inspirent de la proposition de loi de notre collègue Christophe-André Frassa, que le Sénat avait adoptée le 22 janvier 2019. Soucieux d'encourager, au-delà de nos frontières, l'assise démocratique et républicaine des représentants des Français de l'étranger, le RDSE avait approuvé ce texte. Nous avions également soutenu plusieurs dispositions de la loi « Engagement et proximité », relatives à la représentation des Français de l'étranger. Dans la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, nous en retrouvons certaines, parfois satisfaites par la loi du 27 décembre 2019. Par conséquent, en toute logique, mon groupe soutient l'économie générale du titre I, qui pourrait améliorer utilement l'exercice du droit de vote, d'un côté, et l'exercice des mandats, de l'autre. Il s'agirait aussi de favoriser le taux de participation aux élections qui, on le sait, est peu élevé et se trouve même bien en deçà du taux constaté sur le territoire national. C'est une vraie difficulté, pour ne pas dire une fracture démocratique, comme l'avait qualifiée le Président de la République en 2017. Le texte prévoit également des mesures destinées à faciliter la vie quotidienne des citoyens expatriés, notamment en matière de protection sociale et de démarches d'état civil, mesures bien souvent de bon sens. Je souligne ainsi l'intérêt de l'article visant à pallier les conséquences de l'extinction de la compétence notariale des ambassades et consulats. Si la Cour des comptes a réclamé cette évolution, on ne peut pas laisser nos concitoyens sans solution, de surcroît dans les pays qui ne reconnaissent pas l'institution notariale. Le quotidien à l'étranger, c'est aussi celui des enfants des familles expatriées. La question de la capacité des parents à garantir l'accès de leurs enfants au réseau des écoles et lycées français à l'étranger se pose parfois. Je salue à cet égard l'article 19, qui crée une nouvelle catégorie de bourses pour la scolarisation à l'étranger des enfants en situation de handicap. Comme je le soulignais au début de mon propos, la crise sanitaire a affecté l'enseignement, s'agissant notamment de la continuité pédagogique dont certaines familles ont été privées. Le Gouvernement a pris la mesure des difficultés en prévoyant un plan de trésorerie et de revalorisation des aides à la scolarité.

Enfin, nos collègues auteurs de la proposition de loi proposent un volet très important sur la fiscalité, le titre V. Je n'énumérerai pas toutes les mesures que nous avons examinées en commission des finances. Notre collègue rapporteur les a détaillées, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu

Il faut s'extraire d'un tel préjugé puisque les situations sont diverses, allant du modeste retraité au riche. Les propositions doivent répondre à cette hétérogénéité, et c'est ce que la commission des finances a tenté de faire en cherchant des compromis avec les dispositifs initiaux, qui auraient pu favoriser des catégories n'en ayant pas besoin. Pour autant, alors que la France a élaboré l'un des réseaux conventionnels les plus étendus au monde, nous nous retrouvons à réformer la fiscalité des Français de l'étranger, ce véritable « maquis fiscal », pour reprendre l'expression consacrée. Compte tenu de

que des garanties soient apportées sur le respect de l'équité fiscale entre les contribuables français vivant à l'étranger, mais également par rapport aux contribuables hexagonaux. Mes chers collègues, malgré quelques réserves de prudence sur la question fiscale,

Comme dit le chef de l'État, la France protège tous ses enfants. En ce qui concerne le plan des institutions et des élections, le week-end dernier, les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires auraient dû élire leurs élus locaux. Nous ne connaissons pas les nouvelles dates du scrutin, qui seront fixées lorsque le conseil scientifique aura remis son rapport au Gouvernement.

Une seule chose est certaine : les futurs conseillers des Français de l'étranger bénéficieront des avancées prévues par la loi dite « Engagement et proximité ». Grâce à la revalorisation de leur rôle, ils pourront continuer à s'engager et à donner à notre République un visage concret et accessible.

Il convient aussi de rappeler que la loi prévoit l'obligation de motiver les décisions de refus prises contre l'avis des élus, ainsi que l'instauration d'un droit à la formation. Ces points sont importants, car, trop souvent, les propositions votées les propositions votées par les élus sont balayées par l'administration. Enfin, la commission des lois a tiré les conséquences de l'adoption de la loi « Engagement et proximité » en supprimant de la proposition de loi initiale les dispositions dont l'objet est déjà satisfait. Parmi les dispositions d'ordre social, celle qui prévoit l'exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine emporte ma pleine adhésion.

à l'intérieur de l'Union, soit également applicable aux Français qui habitent au Ghana ou à Singapour. Cette solution est plus acceptable que celle, défendue par certains membres de la majorité sénatoriale, qui consistait à exonérer de prélèvements sociaux tous les non-résidents, y compris ceux qui sont à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.

Il n'est pas bon de modifier en permanence la loi ou les décrets qui viennent d'être pris. Je partage également la volonté de nos collègues du groupe Les Républicains de permettre aux retraités ayant cotisé moins de quinze ans de bénéficier d'une prise en charge de santé lors de leur séjour en France.

Pour ce qui concerne les mesures fiscales, je constate que la commission des finances a, dans une certaine mesure, tempéré les ardeurs des auteurs de la proposition de loi. Plusieurs dispositions prévues dans le texte initial, difficilement compatibles avec notre Constitution, ont été remplacées par des mesures que nous avions eu l'occasion de proposer lors de précédents débats.

en revanche, avec la volonté de la majorité sénatoriale d'abroger purement et simplement la réforme de la retenue à la source spécifique aux revenus salariaux. Le dispositif prévu par la loi de finances initiale est loin d'être parfait, et nous avons été nombreux à

d'en discuter et de l'enrichir. Il est difficile d'être défavorable à la suppression du taux minimum d'imposition de 30

nos compatriotes établis à l'étranger est aujourd'hui estimé à près de 3 millions. Je parle bien d'estimation, car nous touchons ici une première difficulté, celle de l'inscription sur le registre des Français établis hors de France. La crise mondiale du Covid-19 a montré, une nouvelle fois, l'importance de cette inscription facultative pour le suivi et l'accompagnement de nos compatriotes par des services consulaires qui n'ont pas ménagé leurs efforts ces derniers mois. Nos compatriotes Nos compatriotes établis à l'étranger ont d'autres problèmes spécifiques. De nombreux expatriés, toujours attachés à la France, ont besoin que l'État français reste présent, notamment dans le cadre démocratique. Je rejoins ici le constat d'une démocratie française à l'étranger en grande difficulté, avec des taux d'abstention record. S'il faut saluer l'opération impressionnante de rapatriement des Français présents à l'étranger, menée par le ministère et les services consulaires depuis le début de la crise du Covid-19, cette action ne doit pas cacher les profondes difficultés que connaissent les services. L'année dernière, plus de 150 demandes de missions de renfort n'ont pu être satisfaites, alors même que le ministère s'appuie de plus en plus sur des recrutés locaux et des contractuels. Il est donc urgent de revenir sur les objectifs fixés par le comité Action publique 2022, qui prévoyait la suppression de nombreux postes.

D'une part, l'objectif poursuivi est de s'appuyer toujours davantage sur les établissements conventionnés et partenaires, ce qui explique en partie le poids toujours plus important des familles dans le financement de l'AEFE.

Monsieur le secrétaire d'État, le plan d'aide que vous avez annoncé le 30 avril était nécessaire pour permettre aux établissements de survivre. Toutefois, sera-t-il suffisant ?

En parallèle, ne devrions-nous pas repenser la relation entre les Français de l'étranger, la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, et la caisse primaire

à leur retour, ils nous rapportent leur dynamisme et une expérience enrichissante et unique : les « expats » participent au rayonnement de notre pays sur le plan économique, culturel, ou linguistique. 206 postes consulaires, chargés de les accompagner dans leurs démarches, font du réseau consulaire français l'un des premiers au monde. Toutefois, nos compatriotes expatriés doivent faire face à des difficultés grandissantes dans leur vie quotidienne. Leur première source d'inquiétude concerne l'éducation et l'accès à l'enseignement du français, malgré le travail de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. En outre, les Français établis hors de France subissent, en raison de leur éloignement géographique, une forme de fracture démocratique, bien qu'ils désirent maintenir des liens avec la communauté nationale. Quant aux démarches administratives, elles sont pour eux d'une grande complexité : je pense notamment aux certificats de vie et aux actes notariaux. Enfin, les questions sociales et fiscales demeurent un enjeu majeur, bien que la France ait signé plus de 120 conventions fiscales afin de réduire les risques de double imposition. Pour répondre aux besoins spécifiques des Français établis hors de France, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui établit un plan transversal couvrant cinq domaines d'action : la représentation politique, les actes notariés, le réseau éducatif, la protection sociale et le régime fiscal. apporte des réponses concrètes à leurs difficultés pratiques et revêt donc une grande importance pour tous les Français de l'étranger. J'en aborderai ici les trois premiers aspects. Tout d'abord, concernant la représentation des Français établis hors de France, la présente proposition de loi vise à améliorer le régime électoral des conseils consulaires consulaires et de l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle s'inspire de l'excellente proposition de loi de notre collègue Christophe-André Frassa, que nous avons examinée et adoptée le 22 janvier 2019. texte sécurise ainsi l'enregistrement des candidatures et l'organisation de la propagande électorale. Il améliore les conditions d'exercice des mandats de conseiller des Français de l'étranger et de membre de l'Assemblée des Français de l'étranger, notamment en ce qui concerne la prise en charge de leurs frais de mandat et leur place dans l'ordre protocolaire. À cet égard, je me réjouis que la commission des lois ait complété le texte, en permettant la prise en compte de l'exercice de ces mandats dans la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes universitaires, ou encore en favorisant l'accès au télétravail pour les élus travaillant dans une entreprise ou une administration française. Ensuite, cette proposition de loi tend à simplifier les démarches administratives des Français à l'étranger. Elle facilite ainsi la rédaction des actes authentiques, évitant de la sorte aux expatriés d'avoir à revenir en France pour se rendre chez un notaire. Ce dispositif a été sécurisé en commission. À titre expérimental, les personnes qui résident hors de France pourraient recourir à des systèmes de visioconférence, l'acte authentique étant établi à distance par un notaire français. Les conditions de délivrance des certificats de vie seraient également simplifiées. Les retraités qui résident hors de France se présenteraient directement à l'ambassade, au consulat ou dans une mairie française.

: 1 295 dans le premier degré et 442 dans le second. Toutefois, certaines familles sont contraintes de scolariser leurs enfants dans des établissements spécialisés extérieurs à l'AEFE et risquent de perdre leurs droits à bourse. Pour répondre à cette difficulté, cette proposition de loi crée une nouvelle catégorie de bourses dédiées au financement des dispositifs de compensation du handicap. Ce dispositif concernerait les établissements de l'AEFE, mais également des établissements tiers, lorsque l'enfant n'aurait pu être accueilli dans le réseau de l'agence. Voilà les principaux éléments qui font que cette proposition de loi illustre l'engagement de notre assemblée en faveur de nos compatriotes expatriés. Je me réjouis que les travaux en commission

un regret : ce texte n'apporte pas de réponse aux difficultés que rencontrent nos compatriotes expatriés à joindre les services publics français depuis leur pays de résidence, malgré l'existence d'un annuaire téléphonique des autorités publiques sur internet : certains numéros demeurent payants et inaccessibles depuis l'étranger.

mes premiers mots iront à M. Retailleau et à ses collègues du groupe Les Républicains, que je tiens à remercier de cette proposition de loi. Son examen nous permet d'évoquer plusieurs sujets intéressant nos compatriotes résidant à l'étranger, ceux-là mêmes que notre ancien collègue Jean-Pierre Cantegrit avait baptisés « la troisième France » dans le livre qu'il leur avait dédié. Au terme de neuf semaines de confinement passées à mon domicile au Royaume-Uni, je veux commencer mon propos en adressant mes pensées chaleureuses et solidaires aux malades du Covid-19 et toute ma compassion aux personnes endeuillées.

Aussi, au moment où je me retrouve dans cet hémicycle, après plus de deux mois de travail à distance, je veux dire à ceux qui sont dans la difficulté que mes pensées sont tournées vers eux.

Les revirements que nous observons sur ce sujet créent un climat anxiogène, nourri d'incertitude administrative et de méfiance sanitaire. Monsieur le secrétaire d'État, pourrez-vous nous rassurer sur cette question ?

des Français de l'étranger n'est pas, à leurs yeux, une réussite. L'expérience montre qu'il faudrait trouver une solution pour que tous les élus consulaires puissent participer activement aux travaux de l'AFE d'une manière ou d'une autre.

ailleurs, le problème principal auquel les élus sont confrontés relève non pas de la loi, mais de son exécution par l'administration. Des témoignages qui me remontent de toutes parts

À titre d'exemple, je veux vous livre ce témoignage : « Je n'ai jamais eu de nouvelles des îlots. Je ne sais même pas qui est chargé de l'îlot dans ma région. À chaque question, je reçois une réponse évasive. Des élus chevronnés notent que la reconnaissance à leur égard se dégrade. L'un m'a ainsi déclaré : « Quand mon pays d'adoption avait connu une révolution, j'avais été associé aux efforts du consulat pour venir en assistance aux Français. Maintenant, c'est fini

cette initiative n'a pas été du goût de l'ambassade de France, qui a empêché le vol en écrivant : « Les étudiants français de Roumanie ne sont pas en situation de détresse, même si leur situation est inconfortable. »

a parfois manqué d'éloges vis-à-vis de nos élus de terrain, dont beaucoup se sont impliqués avec zèle pour aider nos compatriotes bloqués à l'étranger. L'accès aux listes électorales consulaires semble par ailleurs devenir de plus en plus compliqué pour les élus : beaucoup m'ont dit qu'ils n'avaient pu avoir accès aux plus récentes.

J'en connais de nombreux ; je veux les saluer et leur faire part de toute ma gratitude. Nous sommes amenés aujourd'hui à légiférer sur des formalités qui empoisonnent la vie de nos compatriotes et qui devraient être réglées sans même l'intervention du législateur, comme les certificats de vie ou les actes notariés. J'y reviendrai au cours des débats et présenterai trois amendements de ma collègue Nathalie Goulet, inspirés par son travail de lutte contre la fraude sociale.

Hormis quelques articles des lois de finance et de financement de la sécurité sociale, il est vrai que le Sénat examine assez peu souvent des dispositions relatives aux Français de l'étranger. Or, en l'espace d'un peu plus de deux ans,

J'ai bien dit « deux textes » : en effet, s'appuyant sur les travaux de la commission des lois, relatifs au bilan de l'application de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le Sénat a adopté, le 22 janvier 2019, une proposition de loi tendant à améliorer le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France et les conditions d'exercice des mandats électoraux de leurs membres. Cette proposition de loi, adoptée par 327 voix contre 17- nous tenterons de faire encore mieux ce soir

Au lieu de cela, plusieurs dispositions adoptées dans cette proposition de loi se sont retrouvées, comme par magie et, si j'ose dire, quelque peu à l'arraché, dans la loi Engagement et proximité promulguée le 27 décembre dernier. Attendue depuis de nombreuses années, cette avancée reprend en effet la proposition de loi que le Sénat avait adoptée en janvier dernier. Je ne vous ferai pas l'affront, mes chers collègues, de vous rappeler qui en était l'auteur, puisque tout le monde l'a déjà cité ! C'est une grande victoire pour les élus des Français de l'étranger, qui s'investissent partout

Cependant, sur mon initiative, le Parlement a également consacré le droit, pour les conseillers des Français de l'étranger, d'accéder à des formations adaptées à leurs fonctions, comme tous les élus de la République, et a étendu et a étendu les compétences des conseils consulaires, qui seront désormais consultés sur les moyens mis à la disposition des conseillers des Français de l'étranger pour exercer leur mandat. L'ensemble de ces avancées s'appliquera dès les prochaines élections consulaires, dont il ne reste qu'à fixer la date. Il nous faut maintenant aller plus loin. C'est tout l'objectif de la proposition de loi du président Retailleau ; il s'agit aujourd'hui d'apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les Français de l'étranger. Comme il a déjà été rappelé, ce texte, adopté sur le rapport de notre collègue Jacky Deromedi, dont je salue ici le formidable travail, comprend 31 articles couvrant cinq domaines, à savoir la représentation politique, les actes notariés, le réseau éducatif, la protection sociale et le régime fiscal.

tiens à le redire -le fruit d'un important travail, rigoureux, précis et exhaustif, portant sur nos 3,4 millions de compatriotes qui vivent ou qui travaillent hors de nos frontières et qui se voient, depuis plusieurs années maintenant, privés de nombreux droits qu'ils avaient acquis ou que nous avions obtenus pour eux.

Le texte déposé par le président Retailleau et que nous examinons sur le rapport de notre collègue Jacky Deromedi offre des réponses concrètes à autant de questions sur lesquelles nous nous battons depuis de nombreuses années. Cette proposition de loi aura également le mérite de mettre en lumière une collectivité de fait, sinon de droit : celle des Français de l'étranger, qui fait trop souvent l'objet de préjugés. On se focalise souvent sur deux ou trois personnalités résidant à l'étranger, ce qui est par rapport à l'effectif total : en pratique, 65 % des Français de l'étranger paient un impôt à la République à un titre ou à un autre. Aussi, ne serait-ce que pour cette raison, il convient de s'intéresser au « maquis

des problématiques rencontrées par les Français de l'étranger, qu'il s'agisse de leurs instances représentatives- la loi Engagement et proximité a seulement réglé quelques problèmes liés à l'exercice du mandat des élus

Même si je me rallie à l'expérience et à la grande sagesse du président de la commission des lois, qui répondit alors qu'« il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer », il faudra cette fois y veiller, monsieur le secrétaire d'État. Un deuxième acte manqué serait très mal vécu, c'est peu de le dire

Il n'y va pas seulement de la crédibilité du Gouvernement : il y va du respect pour le travail du Sénat et, surtout, du respect dû aux Français de l'étranger, qui se sont, eux aussi, lassés de toutes ces promesses non tenues. La parole

Nous ne sommes évidemment pas dupes : cette initiative prise en mars dernier, avant la crise sanitaire, était d'abord un message envoyé à nos compatriotes établis hors de France, à quelques semaines de la tenue des élections consulaires qui devaient avoir lieu en mai. force est de constater que certains de ses articles, une fois amendés et précisés en commission, se rapprochent nettement de la position défendue par les élus socialistes.

Nous approuvons ainsi le rétablissement des taux de barème progressif antérieurs à la loi de finances pour 2019 ; cela préserverait les Français de l'étranger, notamment ceux dont les revenus sont modestes, d'une hausse brutale

mise à mal par la politique fiscale menée depuis trois ans. Il en est de même du dispositif proposé en matière de crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des logements.

que les plus aisés d'entre eux et ne prend pour exemple que les cadres expatriés. L'éventail des situations sociales est très large, et les Français modestes vivant à l'étranger sont nombreux. L'équité doit donc être notre guide.

cette proposition de loi est très axée sur la propriété immobilière, au risque d'entrer en contradiction avec d'autres objectifs prioritaires des politiques publiques, notamment l'accès au logement de tous dans les

à prendre en compte certains sujets, qui nous paraissent bien plus essentiels, mais qui ne figurent pas dans ce texte, comme les frais induits par la scolarité des enfants à l'étranger ou encore la protection sociale de nos compatriotes. Enfin, comme l'a rappelé M. Retailleau lui-même, nous manquons de données chiffrées pour prendre des décisions suffisamment éclairées. La méconnaissance par l'administration du nombre, des revenus et de la situation fiscale précise des contribuables non résidents limite beaucoup notre vision. En conséquence, le coût global pour les finances publiques de cette proposition de loi reste un mystère, ce qui pose, vous en conviendrez, un vrai problème.

le président Valéry Giscard d'Estaing avait qualifié la France de « grande puissance moyenne

On sait que la crise suscite un certain nombre de défis : baisse potentielle du nombre d'apprenants, interruption des activités culturelles, incertitudes sur les dates et les conditions de réouverture. Nous veillerons toutefois,

vivre la vie démocratique à l'étranger et qui n'ont pu faire encore campagne, on doit dire à quel moment ils pourront le faire. Il est donc urgent, monsieur le secrétaire d'État, de nous dire ce que vous envisagez de faire. Bien entendu, la question des élections sénatoriales On le sait, il est assez peu probable qu'il soit complètement conforme aux exigences du Conseil constitutionnel de réaliser une troisième fois une élection sénatoriale pour les Français de l'étranger avec le même corps électoral, élu en 2014.

dans trois ans ? Il existe plusieurs options, mais on ne peut pas rester dans l'incertitude et on ne peut plus espérer une solution qui vienne d'ailleurs.

Tout le monde s'accorde pourtant sur le fait que ce calendrier n'est pas tenable. Les candidats ne peuvent pas faire campagne, l'administration n'aura pas le temps de contrôler

partage cet avis et recommande de reporter les élections consulaires. Nous attendons donc des réponses de la part du Gouvernement. En tout état de cause, un report des élections consulaires entraînerait le report de l'élection des sénateurs des Français de l'étranger, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Nous devons donc mener une réflexion d'ensemble sur tout ce cycle électoral, en fonction également de ce qui sera décidé pour les élections municipales. En conséquence, nous souhaitons entendre l'avis du Gouvernement.

le corps électoral des sénateurs élus sur le territoire national. Il y a donc plusieurs arbres de possibilités pour les sénateurs établis hors de France.

en situation d'organiser dans les meilleures conditions possible, pour les Français établis hors de France, cette expression démocratique. Il y a des élus, ils sont en poste. Il est vraisemblable désormais qu'il faille de nouveau prolonger

fermé. Quel est l'avis de la commission ? L'inscription reste toutefois facultative, ce qui ne facilite pas le travail de l'administration consulaire. Je suis donc favorable à l'amendement de Mme Goulet, qui rend cette inscription obligatoire. Sa rédaction devra sans doute être précisée à l'occasion de la navette parlementaire, le régime des Français établis hors de France n'étant pas un statut à proprement parler. En outre, je rappelle que l'inscription sur les listes électorales consulaires est un droit pour pouvoir voter. Elle ne peut pas être subordonnée à l'inscription au registre consulaire.

pour les candidats aux élections consulaires. Certains candidats se trouvent très éloignés, souvent de centaines de kilomètres, du chef-lieu de la circonscription électorale. Il leur est difficile de s'y rendre pour faire enregistrer leur

s'agit d'un amendement de repli. Dans les circonscriptions géographiquement étendues comprenant plusieurs pays, il est difficile pour les candidats de se déplacer au chef-lieu afin de déposer leur candidature. L'adoption de cet amendement rendrait possible le dépôt de candidature auprès d'un poste consulaire

Aujourd'hui, les candidats doivent déposer leur candidature auprès de l'ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Cela pose des difficultés pour les Français de l'étranger, car les circonscriptions peuvent être particulièrement étendues, notamment pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Je suis donc favorable à l'idée de simplifier les procédures. À l'avenir, il faudra peut-être envisager un dépôt de candidature dématérialisé, ce qui nécessitera de nouveaux développements informatiques de la part du consulat. Les dispositions de l'amendement n° 29 rectifié me semblent constituer un bon compromis. Elles permettent de déposer la déclaration de candidature dans toute ambassade ou tout consulat de la circonscription.

La crise sanitaire nous oblige à adapter nos processus électoraux, en particulier pour les élections des Français de l'étranger. Quelle que soit la date des prochaines élections, il sera difficile, voire impossible, d'accéder aux bureaux de vote qui se situent parfois à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile. Il existe certes le vote par internet, mais plus d'un quart des électeurs inscrits n'a pas transmis son adresse électronique. Les auteurs de l'amendement n° 27 rectifié proposent donc à ajouter la possibilité de voter par correspondance papier. Ils se limitent d'ailleurs à reprendre le droit applicable aux élections législatives.

Je partage entièrement ce qui vient d'être dit. Je ne connais pas beaucoup de régions, même au fin fond de l'Afrique, où il n'y ait pas d'accès à internet-

en délégués électoraux, pour éviter toute confusion. En effet, l'unique rôle des délégués consulaires est de participer, tous les trois ans, à l'élection des sénateurs des Français de l'étranger. La dénomination de délégué électoral nous semble donc plus appropriée à la fonction. De plus, elle éviterait une confusion, parfois savamment entretenue.

délégués consulaires ont bien pour fonction de voter aux élections sénatoriales, ils sont également les suppléants des conseillers consulaires en cas d'épuisement de liste. Changer leur titre ne modifierait pas leurs fonctions. L'avis de

puisqu'ils ont d'autres fonctions que de participer à l'élection des sénateurs. Mais

est à M. Jean-Yves Leconte. L'article 12 apporte de nouvelles garanties aux conseillers des Français de l'étranger et aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'exercice de leurs mandats. Il est notamment prévu que ces élus bénéficieront d'autorisations d'absence pour assister aux réunions liées à l'exercice de leur mandat. Malheureusement, ces dispositions, qui vont dans le bon sens, ne s'appliqueront qu'aux employeurs relevant du droit français. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à poser le principe, applicable à tous, employés d'une entreprise ou d'une administration française et employés d'une entreprise ou d'une administration étrangère,

La commission des lois a substantiellement renforcé les droits des élus des Français de l'étranger, notamment lorsque ceux-ci doivent assister aux réunions des conseillers consulaires. Les dispositions de l'amendement n° 20 s'inscrivent dans la même logique, en prévoyant que, d'une manière générale, la convocation aux réunions tient compte des obligations professionnelles des conseillers des Français de l'étranger. La mise en oeuvre de ce dispositif sera d'autant plus facile que la présidence des conseils consulaires sera prochainement exercée par un membre élu. L'avis de la commission est donc favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Les conseillers consulaires sont les élus locaux des Français de l'étranger et perçoivent à ce titre des indemnités, calculées sur la base d'une indemnité mensuelle de référence d'un conseiller municipal d'une ville de moins de 100 000 habitants, majorée au titre de l'expatriation, à laquelle s'applique un indice de base dit « indice Mercer », permettant de tenir compte des disparités du coût de la vie dans les différents pays. Ce calcul ne prend aucunement en compte la dimension de la circonscription que les conseillers consulaires ont à couvrir- parfois plusieurs pays -, ni la taille de la communauté française qu'ils ont à représenter,

tend à soulever une question importante, relative aux indemnités de fonction des conseillers consulaires : dans quelle mesure pourrions-nous moduler cette indemnité en fonction de la taille géographique de la circonscription ? Le droit en vigueur prend en compte le coût de la vie, mais est-ce suffisant ? Je rappelle que certains frais de déplacement sont remboursés, lorsqu'ils sont supérieurs à 60 % de l'indemnité de mandat. En outre, la proposition de loi prévoit déjà des avancées considérables pour que les conseillers consulaires ne soient pas contraints d'avancer leurs frais de déplacement. Ils pourraient ainsi bénéficier d'une avance sur frais de mandat.

Le fonds de soutien au tissu associatif des Français de l'étranger, le Stafe, a été créé en 2018 en remplacement de la de la réserve parlementaire. Doté désormais d'un peu moins de 2 millions d'euros, il permet de financer des projets associatifs de nature caritative, culturelle, éducative ou socio-économique.

La répartition des aides est actée par des commissions locales, puis par une commission nationale, qui procède aux arbitrages. Présidée par la directrice des Français de l'étranger et de l'administration consulaire, la commission compte des membres de l'administration, ainsi que des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger et des associations représentatives de nos compatriotes expatriés. Cet amendement vise à compléter la composition de la commission nationale, en y ajoutant un député et un sénateur

Le fonds Stafe, qui a été créé en 2018 pour soutenir les projets associatifs, occupe une place croissante, même si son montant reste limité à 2 millions d'euros. L'adoption de cet amendement permettrait deux avancées majeures : d'une part, clarifier le fonctionnement de la commission chargée de répartir ces financements,

de l'étranger hors de l'espace Schengen. Vous ne pouvez pas imaginer la confusion et les inquiétudes que ces dispositions ont

Les Français de l'étranger s'inquiètent beaucoup de l'obligation de quarantaine qui pourrait leur être imposée à leur retour sur le territoire national, alors qu'ils subissent dans leur pays d'accueil des quarantaines souvent très strictes- elles le sont parfois plus Lors de l'examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, nous avions proposé de soumettre cette quarantaine à l'existence d'un test positif. Cela n'a toutefois pas été possible à cause du manque de fiabilité de ces tests, comme l'avait souligné le président Bas. Cet amendement vise à prendre acte de cette impossibilité. Ses auteurs prévoient toutefois plus de transparence, en demandant au ministre de la santé d'actualiser au moins chaque semaine la liste des pays considérés comme à risque. La liste de ces pays serait également publiée sur le site des ambassades et des consulats- une semaine après l'adoption de la loi du 11 mai, j'avoue ne pas avoir trouvé cette liste, monsieur le secrétaire d'État

dans leur pays de résidence. Le travail consécutif à l'adoption de la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire est en cours. Il est même en passe de s'achever,

d'un espace géographique comprenant des pays où la circulation du virus est intense. D'un point de vue sanitaire, cela n'avait absolument aucune logique,